Je suis fort surpris de l'évacuation par la commission spéciale de nombreux amendements déposés. Je rejoins mon collègue Fabien Gay, qui s'étonnait en début d'après-midi du sort réservé à de nombreux amendements, déclarés irrecevables comme cavaliers.

ouvrirait la possibilité à ce terroir de produire et de commercialiser la clairette rosée, produit qui n'existait pas en 1957, car il ne correspondait pas alors aux goûts des consommateurs. Aujourd'hui, ce besoin existe, mais ce créneau est occupé par les vins effervescents espagnols et italiens, qui envahissent le marché et font concurrence à un savoir-faire de nos territoires. On ne peut produire ce vin qui permettrait des débouchés intéressants à l'appellation, alors que des possibilités de réviser cette loi existaient à travers ce texte. Je le regrette vivement. Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue. La parole est à

une mission de caractère public et d'un intérêt majeur. Certes, il ne s'agit pas de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Toutefois, derrière la réforme proposée, le premier objectif, ne nous y trompons pas, est encore et toujours de réaliser une économie budgétaire. Mais vous n'avez pas misé sur la nécessaire stabilité financière dont devrait disposer le réseau des CCI ni sur un dialogue renouvelé avec les partenaires du terrain. Vous avez au contraire ouvert une brèche conduisant à la privatisation du réseau. En détournant les CCI de leur mission de service public, vous les réorientez vers des prestations payantes aux entreprises, ce qui les transformera en quasi-cabinets de conseil, à la main de ceux qui en auront les moyens. Ce qui était un service public à destination du milieu économique va se transformer désormais en prestations payantes. En effet, effet, lorsque le conseil consulaire recule, il n'est pas remplacé par un conseil public provenant du département, de la région ou de la communauté de communes : il est remplacé par un service privé. Cela peut être très discriminant et relaie rarement les préoccupations éthiques que portent par essence les chambres consulaires, lesquelles sont détentrices d'un mandat de la République et relèvent de fonds publics et d'une éthique collective. C'est une dénaturation profonde de ce réseau à caractère public à laquelle nous nous opposons fermement.

partout et seulement à des prestations de services numériques. Nous souhaitons ainsi donner la possibilité aux nouvelles organisations de s'adapter plus finement aux conditions techniques, économiques et culturelles d'accès aux prestations proposées. Il ne peut y avoir un seul modèle de services proposé. Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il serait utile de prévoir, dans un premier temps au moins, des guichets téléphoniques et des accueils adaptés pour celles et ceux qui n'utilisent pas ces prestations numériques.

La transformation ici proposée n'est en aucun cas un gage d'efficacité dans l'exercice des missions des CCI, bien au contraire. Relevant d'une idéologie dépassée, qui considère que fragiliser les conditions de travail et remettre en cause des statuts rime avec efficacité économique, la mesure contenue dans cet article n'a pas lieu d'être mise en place. Aujourd'hui, 20 000 agents employés dans les CCI bénéficient d'un statut d'agent public. Un peu moins de 3 000 personnes travaillent quant à elles dans des équipements gérés par les CCI et sont soumises à un statut de droit privé. Vous nous dites que cela est source de complexité. Pourquoi alors ne pas simplement étendre le statut d'agent public à toutes les personnes qui travaillent dans et pour les CCI ? Un autre argument- qui devient une habitude -consiste à dire que ces agents publics bénéficient d'indemnités de licenciement très supérieures à celles qui sont prévues par le code du travail. Vous prétendez que cela n'est pas bon pour les personnels. Nous ne partageons pas ce point de vue et les jugements récents de conseils de prud'hommes nous donnent raison. Vous avez l'objectif de remplacer des agents de terrain qui connaissent bien le tissu économique, qui travaillent dans la durée avec les entreprises et qui sont spécialisés dans des domaines liés à l'activité économique de leur territoire, par des personnes disposant de contrats de mission. viendront pour un contrat de six mois, voire d'un an, en ayant pour mission de dynamiser une activité ou d'accompagner un plan de développement économique élaboré en liaison avec les régions. Cela ne marchera pas, car il faut un personnel de proximité qui connaisse le territoire, qui ait un lien direct avec lui. Au final, tout ce mécanisme n'est qu'un habillage pour justifier des réductions de dépense publique. L'amendement Cet amendement vise à modifier les dispositions de la convention collective relative aux personnels des CCI afin de garantir la possibilité d'adaptations au niveau régional, dans le cadre des CCI de région. Ainsi, les personnels des chambres seront régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France et les organisations syndicales représentatives au niveau national. CCI France animera et présidera l'institution représentative nationale du réseau. Elle négociera et signera les accords collectifs nationaux en matière sociale. Ces accords seront applicables aux personnels des chambres, y compris dans les domaines relevant de la négociation collective de branche,

Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, le projet de loi PACTE habilite le président de CCI France à conclure la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé des CCI à compter de la date de son agrément. En l'état actuel, ce dispositif restreint sensiblement les champs de négociation de chaque CCIR employeur à ceux qui sont autorisés par la convention collective nationale, ne laissant aucune souplesse possible et empêchant ainsi les CCIR employeurs de déroger aux dispositions y figurant, même de façon plus favorable. La mise en oeuvre d'un tel dispositif engendrerait en outre des risques contentieux importants, en empêchant certaines CCIR d'utiliser le droit qu'elles tirent de la loi de mettre en place un dispositif d'épargne salariale et de retraite supplémentaire à cotisations définies. L'objet de cet amendement est donc de définir dans la loi les domaines d'intervention et les conditions d'application de la convention collective nationale en référence aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, qui fixent le contenu des conventions de branche et l'articulation avec les normes inférieures. Une telle disposition permettra aux CCI employeurs de bénéficier de tous les avantages d'une convention de branche sans avoir à en créer une nouvelle, tout en laissant la possibilité de garantir et de préserver les situations spécifiques des CCI employeurs dans la convention collective nationale.

les personnels concernés qui refuseraient le contrat ou l'engagement qui leur est proposé par le repreneur de cette activité se verraient appliquer les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail qu'ils tiennent du statut administratif qui leur est applicable. Il apparaît en effet complexe juridiquement de faire appliquer par les entités d'accueil aux agents publics concernés des mesures relevant d'autres dispositions que celles prévues par le statut des chambres. L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Capus,

vise à maintenir et à favoriser le dialogue social au niveau des CCI de région, en cohérence avec le régime appliqué aux entreprises de droit privé, tout en confirmant le rôle de tête de réseau de CCI France, qui animerait la branche et la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation prévue par le code du travail.

n° 957 vise à modifier les dispositions relatives au transfert des prérogatives des instances représentatives des personnels des CCI afin de garantir le fait que les prérogatives jusqu'alors exercées par les commissions paritaires régionales des établissements du réseau et par la commission paritaire de CCI France seront exercées par les institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau, en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

ne pouvait pas répondre aux aspirations des Français. Il l'a pourtant fait pendant des années, notamment depuis que le général de Gaulle nationalisa un certain nombre d'entreprises, ce dont nous nous félicitons encore aujourd'hui.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Cet amendement vise à rendre possible l'union volontaire d'une ou de plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales à une CCI métropolitaine, sans dissoudre totalement les établissements publics concernés. les établissements publics concernés. Seules les CCI territoriales seraient dissoutes, la CCI métropolitaine recevant la dévolution des droits et obligations des CCI territoriales dissoutes et étendant sa circonscription aux circonscriptions de ces dernières. L'objectif est de reproduire, sur la dimension métropolitaine, le schéma adopté pour l'union d'une CCI territoriale à la CCI régionale. s'en trouverait ainsi facilité et serait plus rapide que la dissolution-dévolution actuellement prévue entre les CCI territoriales, y compris métropolitaines, et utilisée pour la création juridique des CCI Alsace Eurométropole et Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

Cette faculté s'ajouterait à celle déjà prévue par le code de commerce permettant à des CCI territoriales de s'unir à leur CCI de région. Il faut rappeler que les chambres métropolitaines sont juridiquement des CCI territoriales. Si elles sont qualifiées de métropolitaines, c'est parce qu'elles se situent dans le ressort d'une métropole.

aux découpages tels qu'ils existent, pour être plus efficaces au service de l'activité économique de nos territoires.

Peut-être aurai-je plus de succès avec cet amendement ... Votée avant la loi MAPTAM et la loi NOTRe, la loi du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire n'a pas traduit le fait métropolitain dans l'organisation consulaire. une dénomination de chambre métropolitaine sans que les compétences de l'établissement public en soient modifiées par rapport à la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le dispositif proposé par cet amendement consiste à introduire dans la loi des des compétences étendues des CCI métropolitaines, notamment par la voie conventionnelle, relatives à l'animation économique spécifique de l'aire métropolitaine, compétences dépassant celles des CCI territoriales et adaptées à l'aire d'une métropole. L'amendement vise aussi à préserver la personnalité morale des CCI métropolitaines dans le cadre du processus de rapprochement et de mutualisation des chambres de commerce et d'industrie du réseau, compte tenu des spécificités énoncées ci-dessus et de la mise en cohérence avec la loi MAPTAM.

son articulation n'est pas assurée avec les dispositions de l'article L. 711-1 du même code, qui prévoit qu'une CCI territoriale peut déjà prendre la dénomination de CCI métropolitaine et être désignée comme agence économique de la métropole.

J'ai du mal à accepter l'idée que la Nation se divise en une série d'entités particulières qui ne se mélangent pas. C'est pourquoi l'idée de métropole me gêne

la seconde ayant tendance à vivre sur elle-même, à s'enfermer dans ses richesses et à profiter de l'ensemble des moyens dont elle dispose en oubliant qu'il y a aussi une périphérie à faire vivre.

Martine Berthet. Le présent projet de loi prévoit de donner plus de pouvoirs à CCI France. Si ces mesures peuvent permettre une meilleure harmonisation des stratégies consulaires régionales avec l'ensemble du territoire national, il paraît indispensable de renforcer le processus démocratique de cette institution- les membres de son assemblée générale ne disposent aujourd'hui que de très peu de pouvoirs. C'est pourquoi cet amendement ouvre la possibilité pour l'assemblée générale de CCI France d'amender les décisions proposées par le président et son comité directeur

permet déjà la collégialité. En effet, un comité directeur composé du président de CCI France, de tous les présidents de CCI de région et des présidents de CCI membres du bureau

Il nous semble que le fonctionnement de CCI France est plutôt un modèle de démocratie participative, qui ne justifie pas de préciser que les présidents de CCI ont un droit de censure sur les décisions

Le présent amendement vise à limiter à soixante-cinq ans l'âge à partir duquel ne peut plus être élu un président de chambre. Il s'agit d'ajouter une règle spéciale au droit en vigueur.

loi a précisé que la délivrance de ces cartes était confiée aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France. Or, ces dernières étant dépourvues de la personnalité morale, la compétence doit, en toute rigueur, incomber au président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Il en va de même pour les chambres de commerce et d'industrie locales créées depuis 2016, qui sont huit à ce jour, une en Rhône-Alpes et sept dans les Hauts-de-France. Il semble donc nécessaire de préciser que, dans ces circonscriptions, la compétence incombe au président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Quel est l'avis de la commission spéciale ? Cet amendement de cohérence juridique, qui est lié à la restructuration du réseau des CCI et à l'absence de personnalité juridique des chambres départementales d'Île-de-France et des chambres de commerce et d'industrie locales, est tout à fait pertinent. L'avis est donc favorable. Quel est

De fait, le baccalauréat ou une équivalence de niveau est indispensable pour s'inscrire au diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur. Être bachelier apparaît donc comme un frein pour une partie des jeunes voulant s'inscrire dans une démarche entrepreneuriale. C'est pourquoi le présent amendement vise à permettre aux étudiants et aux jeunes diplômés

qui siègent au sein des chambres régionales ne soient pas désignés par un scrutin de liste à la proportionnelle, de donner des moyens

amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l'organisation administrative du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat autour d'un établissement régional, en précisant les moyens d'action des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres départementales, qui doivent être maintenues et renforcées, agiront grâce à un budget d'initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chaque département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire. L'organisation est prévue dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.

12 décembre 2018. Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme, selon leur souhait, devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région du Grand Est, qui entame dès janvier 2019 le processus de régionalisation.

prendrait plus en compte les spécificités du monde des métiers et de l'artisanat. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres collègues de différents groupes, j'ai présenté cet amendement. Il s'agit de respecter la position

date du début de la constitution du réseau uniquement en chambres de métiers et de l'artisanat de région, et octobre 2021, date du renouvellement général de ces chambres. Il

Je vais tenter de vous résumer la situation ... Je vous rappelle que l'article 13 A prévoyait la transformation obligatoire des chambres régionales en chambres de région constituant un seul établissement public par région et dotées de délégations départementales dépourvues de personnalité juridique. La commission a préféré supprimer purement et simplement cet article afin de conserver le choix entre le modèle intégré des chambres de région et celui des chambres régionales, où subsistent des établissements publics départementaux.

Tous ont repris la rédaction que j'avais proposée afin que cette organisation ne remette pas en cause les actions de proximité dans les territoires. Évidemment, je m'en félicite. Certains prévoient d'accorder aux émanations de la CMA de région un budget d'initiative locale. D'autres proposent de renommer les délégations de la chambre de région « chambres de niveau départemental », sans cependant modifier le fait que ces délégations ou chambres restent dépourvues de toute personnalité morale et d'autonomie juridique réelle. encore proposent de nouvelles conditions d'élection des membres des CMA de région et un aménagement de leurs prérogatives. Enfin, un sous-amendement prévoit des dispositifs transitoires pour prendre en considération les prochaines élections des CMA, qui La commission a pris acte de ce renversement de situation et, puisqu'une majorité semble se dégager pour une régionalisation forcée, elle propose de retenir finalement le modèle unique de la CMA de région, avec des chambres départementales dénuées de personnalité morale, mais qui seraient dotées de budgets d'initiative locale et qui mèneraient, pour le compte de la CMA de région, des actions de proximité. Ce dispositif serait complété par les mesures transitoires que j'ai citées.

Simplement, les chemins que nous devrions ou aimerions emprunter sont différents.

Je ne suis intervenu à aucun moment pour interrompre quelqu'un

et de délégations départementales. Je pense, comme ma collègue Monique Lubin, qu'il faut arrêter de vider nos départements des services de proximité en général, afin qu'ils restent vivants. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat fonctionnent très bien. Celle d'Occitanie est

Permettez-moi de mentionner quelques chiffres. La CMA de PACA a accompagné 15 000 porteurs de projets, soutenu 6 200 entreprises artisanales et 4 500 artisans et revitalise les formalités de 43 000 chefs d'entreprise. Elle oriente par ailleurs 9 500 jeunes, forme 6 000 apprentis et 18 000 chefs d'entreprise. Elle diffuse de l'information auprès de 60 000 entreprises. Autant dire que la structure actuelle fonctionne bien. Pourtant, ce texte souhaite la supprimer. Faut-il appliquer le même modèle d'organisation partout

qui vont adopter ce modèle, choisi à une très forte majorité par les présidents de CMA départementales. Dans la réforme dont nous parlons, les présidents départementaux participeront à la gouvernance de la région, avec une représentation exceptionnelle : un département, une voix. Je pense que l'on ne peut pas faire mieux pour la départementalisation de ce projet. La parole

L'amendement sur lequel nous sommes en train d'échanger consiste à dire que nous conservons des entités départementales. Tous les amendements sur lesquels Mme la rapporteur et Mme la secrétaire d'État ont donné un avis favorable reprennent cette idée.

tous les ans ou à chaque renouvellement des actions communes. Elles le font au fil du temps, en fonction de l'intérêt de leur territoire et de leurs ressortissants. Jouons l'efficacité ! Faisons confiance à ceux qui sont sur le terrain, aux femmes et aux hommes qui ont été élus pour cela.

On a bien vu qu'il y avait une complémentarité entre les chambres consulaires, donc le monde économique, et les collectivités locales, qu'elles soient départementales, régionales, communales ou intercommunales.

On n'imagine pas qu'elles soient suffisamment responsables et compétentes pour décider, entre elles, de la manière dont elles doivent s'organiser. Tous nos territoires sont différents, nos représentations sont différentes, nos configurations géographiques sont différentes ! Ne peut-on pas arrêter de vouloir faire le bonheur des gens contre leur

Cela signifie qu'il peut y avoir un futur aléatoire. Je ne suis pas encore sûr qu'il soit nécessaire de légiférer sur le futur aléatoire.

lisez simplement la rédaction que nous proposons à l'amendement n° 958 : « Dans l'exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat mènent des actions de mutualisation de certains de leurs moyens matériels et d'une partie de leur offre de services ».

aux CMA, aux CCI et aux chambres d'agriculture de discuter en début de mandat de ce qui pourrait être partagé et mutualisé entre elles. C'est simplement une possibilité. Le fait de le préciser dans la loi amène à poser la réflexion,

pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté : comme M. le ministre Bruno Le Maire l'a déjà dit de manière très nette et à plusieurs reprises, tant dans cet hémicycle qu'à l'Assemblée nationale, il n'est pas question de fusionner les CCI et les CMA,

de service unifiée et de centraliser les fonctions support suivantes : opérations d'envergure nationale, programmes informatiques, veille et support juridiques, consolidation budgétaire.

Actuellement, un membre d'une CMA peut exercer sans limitation dans le temps la présidence d'une chambre. Cette absence d'encadrement du nombre de mandats peut nuire à la gouvernance des organismes, voire bloquer toute initiative en faveur d'une modernisation des réseaux consulaires. Il est proposé de limiter ce nombre à deux mandats, soit dix ans, pour toutes chambres confondues. Il s'agit d'impulser un nouveau dynamisme dans le réseau. Cette disposition permettra un renouvellement des organes dirigeants et favorisera l'engagement d'un plus grand nombre de chefs d'entreprise. Quel

Georges Patient. L'Assemblée nationale a adopté un amendement limitant le cumul dans le temps des mandats de président de CCI, quels que soient ces mandats et quelle qu'en soit la durée. Or certains mandats peuvent être très courts- un ou deux mois -lorsqu'ils sont un préalable à l'élection au niveau supérieur, notamment pour les présidences de CCIR ou de CCI France. Cet amendement vise donc à privilégier une approche fondée sur le nombre d'années d'exercice de mandats, correspondant à trois mandats pleins ; le décompte débuterait au prochain renouvellement général. En outre, pour éviter toute rupture en cours de mandat, un membre qui viendrait à atteindre sa quinzième année de mandat de président de CCI en cours de mandature

par décret, de plusieurs CCI territoriales d'une même région qui ne seraient pas en mesure de redresser leur situation financière. Pour défendre cet amendement de suppression, je reprendrai simplement les éléments du rapport de la commission spéciale, qui sont sans appel Cette transformation serait imposée unilatéralement par l'autorité de tutelle et n'interviendrait que lorsque celle-ci a constaté l'impossibilité du redressement de la situation financière des chambres concernées. Or, dans le même temps, il est prévu une baisse de 300 millions d'euros de leur financement public issu de la taxe pour frais de chambre. Dès lors, cet article est une conséquence de la politique de réduction du financement public des CCI. a choisi de mettre en difficulté certains établissements publics infrarégionaux du réseau, qui seront dans une situation financière telle qu'ils ne pourront plus assurer leurs missions. Ainsi, la mise en oeuvre de ce dispositif pourra conduire à la création d'une organisation du réseau des CCI au niveau régional autour d'un établissement public unique- la CCIR -doté de chambres locales dénuées de personnalité et d'autonomie juridiques, le cas échéant contre la volonté des élus de la CCIR. Tout comme la commission spéciale, nous regrettons que les choix financiers du Gouvernement, confirmés par la loi de finances pour 2019 malgré l'opposition résolue du Sénat,

spéciale ? Nous nous sommes régulièrement opposés ces dernières années aux coupes drastiques du financement public dont les CCI ont fait l'objet. puisqu'elles ont été mises dans cette situation, il faut trouver un moyen de préserver leur capacité d'action. Cet article y contribue. Notre commission a par ailleurs conforté juridiquement ces mesures. Elle est donc évidemment défavorable à cet amendement de suppression de l'article.

de directives européennes en droit français, dont j'avais l'honneur d'être le rapporteur pour la commission spéciale, avec ma collègue Martha de Cidrac. Ces dispositions ont pour objet de relever les seuils de définition de la catégorie des petites entreprises au niveau maximal autorisé par le droit européen, en levant une option prévue par la directive dite « comptable que d'étendre aux micro-entreprises et aux petites entreprises qui sont soumises au contrôle des comptes, ou qui s'y soumettraient volontairement, le bénéfice des modalités de publication allégée du rapport des commissaires aux comptes. Dans la mesure où ce projet de loi dit de « dé-sur-transposition » n'a toujours pas été examiné par l'Assemblée nationale- je rappelle qu'on nous avait son examen à toute vitesse ! -, je ne peux que soutenir l'introduction dans le projet de loi PACTE de ces mesures d'allégement et de simplification en faveur des entreprises que j'ai moi-même proposées, afin qu'elles entrent au plus vite en vigueur. Je

Ce concept, relativement récent, mérite quand même quelques observations. Cela voudrait dire que, contrairement à une légende savamment entretenue, les directives européennes ne constituent aucunement le fin du fin et l'étape ultime du droit positif dans notre pays, mais simplement le socle dont il doit être constitué au minimum. Les dispositions incriminées ne sont en réalité et en dernière instance que celles qui peuvent procéder du droit national, de son histoire et de sa construction. À la vérité, quand nous sommes confrontés à une supposée « sur-transposition », c'est tout simplement parce que notre droit positif est bien plus précis et plus avancé que ce qu'exige le minimum européen. Nous pouvions très bien dispenser les entreprises de la publicité de leurs comptes annuels sans contrevenir le moins du monde à la directive. La France, d'ailleurs, plutôt que de se conformer à une règle sans doute demandée et portée par les milieux patronaux européens et relayée, comme il se doit, par le MEDEF, aurait mieux fait, soit dit en passant, d'en appeler à une plus grande transparence, puisque la connaissance que nous aurons demain de notre tissu économique sera plus qu'imparfaite pour le citoyen et ne devra sa précision

M. Cadic me contredira si j'ai tort - : elle compte moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 43 millions d'euros en total de bilan.

il est nécessaire de prendre en compte le principe de continuité du service public, qui implique de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption. Or l'état contrasté de la couverture numérique et l'éloignement géographique de ces structures administratives doivent constituer des critères pertinents pour adapter les moyens mis à disposition pour garantir cette continuité. Ensuite, il paraît nécessaire de conforter le principe d'égalité devant ces missions de service public. À ce titre, des entreprises se trouvant dans une situation identique à l'égard des chambres consulaires doivent être régies par les mêmes règles. Or un territoire constitué par de grandes PME n'est pas le même qu'un territoire constitué d'une plus grande part de TPE : les besoins, les capacités logistiques, mais aussi les chiffres d'affaires ne sont pas les mêmes. Aussi, nous proposons d'inscrire dans le texte des garanties supplémentaires pour que toutes les entreprises, y compris les plus petites d'entre elles, puissent bénéficier d'un accès normal au regard des contraintes géographiques, techniques ou des spécificités économiques dans lesquelles elles évoluent. Quel est l'avis de la commission

pour les chambres de commerce et d'industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année à la majorité simple des membres présents ou représentés à l'assemblée générale de CCI France.

visant à permettre à CCI France de donner un avis motivé et préalable à la nomination de chaque directeur général du réseau. Cet avis simple paraît nécessaire à l'intégration de CCI France dans un processus de recrutement des directeurs, en vue de créer une communauté managériale indispensable à la mise en place d'un véritable réseau. Bien entendu, la décision finale sur le recrutement demeure celle de la CCI employeur.

et de nomination des directeurs généraux des CCI territoriales et de région, ce qui s'inscrit pleinement dans la logique de renforcement du rôle de tête de réseau de CCI France.

on ne choisit pas forcément de manière descendante les uns et les autres. La qualité du, c'est aussi de faire travailler des gens différents, avec des objectifs

la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année à la majorité simple des membres présents ou représentés

: ce sont des institutions ! La relation de confiance qui existe est induite par la proximité : ce sont des relations parfois personnelles qui permettent de débloquer des dossiers ou d'en accélérer d'autres. Ne nous privons pas de ces leviers, surtout dans nos territoires

Mme Corinne Imbert. Cet amendement vise à permettre le financement des CCI territoriales en supprimant l'obligation de fusion lorsqu'elles sont plusieurs dans un même département. En effet, sur certains territoires, il peut y avoir des bassins économiques différents, ayant chacun une taille critique suffisante et assumant la gestion d'équipements structurants, tels que des ports ou des aéroports, pour coexister. C'est notamment le cas du département des Pyrénées-Atlantiques, qui compte un bassin économique autour de Pau-Béarn et un autre autour de Bayonne-Pays basque. Cette disposition, supprimée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 au motif qu'elle constituait un cavalier législatif, a été réintroduite à l'Assemblée nationale. Je ne fais que répéter ce que mon collègue Max Brisson déclarait au mois de décembre dernier, lorsqu'il évoquait les réalités du bassin économique sur lesquelles sont fondées ces CCI. un bassin de 300 000 habitants, la CCI gère un port de commerce, ce qui explique d'ailleurs sa fondation au XVIII siècle, un port de pêche, une école d'ingénieurs réputée qu'elle a créée, ce qui permet une véritable reconnaissance par les entreprises comme par les collectivités. Au moment où la question des territoires, de la proximité, de l'accompagnement au plus près se pose dans le pays, clarifions nos positions en ne laissant aucune ambiguïté sur la pérennité de ces CCI qui fonctionnent, car elles sont en phase avec leur territoire. Quel est l'avis de la commission

Les syndicats mixtes dits « ouverts » sont des établissements publics pouvant être constitués par accord entre des collectivités territoriales, leurs groupements et d'autres personnes morales de droit public, tels que les Le retrait d'un membre, à défaut de dispositions particulières prévues dans les statuts du syndicat mixte, fait l'objet d'une décision prise à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, ce qui peut entraîner des situations où un membre se retrouve contraint de maintenir sa participation contre son gré. Compte tenu des évolutions des missions des CCI et de leur financement opérées par le présent projet de loi, il paraît nécessaire de prévoir un mode de retrait particulier pour les

Mme la secrétaire d'État. Les dispositions prévues à l'article 13 permettront aux CCI employeurs d'adhérer au régime d'assurance chômage pour l'ensemble de leurs collaborateurs, à titre irrévocable, sachant qu'elles seront autorisées à recruter des personnels de droit privé à compter de la publication du présent Pour compenser à l'UNEDIC la charge financière nouvelle créée par cet amendement, notamment concernant l'indemnisation par le régime d'assurance chômage de personnels statutaires appartenant à des établissements publics administratifs de l'État, il est prévu une surcotisation

n'est pas déjà le cas.

de façon contrainte, forcenée, les moyens des CCI, qui vont inévitablement être obligées de recourir à des licenciements. Et là, gentiment, le Gouvernement,

qui prévoit déjà une compatibilité de la stratégie de la chambre de commerce et d'industrie de région avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit ainsi de supprimer l'ajout du mot « complémentaire » dans une phrase qui contient déjà le terme « compatible ». Il paraît en effet conforme à l'objectif recherché par la commission spéciale du Sénat, qui a supprimé l'obligation de conventionner entre les régions et les chambres de commerce et d'industrie, en rappelant que ces acteurs opéraient déjà de tels rapprochements, sans obligation légale.

on souhaite ajouter les mots « complémentaires de celle de la région ». Or, comme cela a été précisé, le code de commerce prévoit déjà des stratégies compatibles entre les CCI et les régions. Il s'agit donc à notre sens d'un degré d'opposabilité suffisamment